est ouverte. Le compte rendu intégral de la séance du mercredi 3 mars 2021 a été publié sur le site internet du Sénat. Il n'y a pas d'observation Le procès-verbal est adopté. J'informe le Sénat que la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi améliorant l'efficacité de la justice de proximité et de la réponse pénale est parvenue à l'adoption d'un texte commun. Par lettre en date du jeudi 4 mars M. François Patriat, président du groupe RDPI, a demandé de réduire à quarante-cinq minutes la durée de la discussion générale sur la proposition de loi rénovant la gouvernance du service public d'eau potable et d'assainissement en Guadeloupe et sur la proposition de loi créant la fonction de directrice ou de directeur d'école, examinées au sein de l'espace réservé à son groupe du mercredi 10 mars 2021. Y a-t-il des observations ? ? ... Il en est ainsi décidé. L'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi tendant à garantir le droit au respect de la dignité en détention, présentée par M. François-Noël Buffet La procédure accélérée a été engagée sur ce texte. Dans la discussion générale, la parole est à M. François-Noël Buffet, auteur de la proposition de loi. Monsieur

Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, le texte qui est aujourd'hui soumis au Sénat, cosigné par des membres de la commission des lois émanant de plusieurs groupes,

la Cour de cassation et le Conseil constitutionnel ont en effet constaté que la loi française ne comportait pas de voie de recours juridictionnel permettant de mettre fin à des conditions de détention indignes en prison. voie de recours. Au mois de janvier 2020, la Cour européenne des droits de l'homme, condamnant la France à indemniser trente-deux personnes incarcérées en métropole et outre-mer pour traitements inhumains et dégradants en application de l'article 3 de la Convention, a pour la première fois jugé que les requérants ne disposaient pas d'une voie de recours effective pour faire cesser ces conditions de détention indignes. Cela constitue une violation de l'article 13 de la Convention, qui reconnaît à toute personne dont les droits et libertés ont été violés le droit à un recours effectif devant une instance nationale. de juillet 2020, la chambre criminelle de la Cour de cassation a tiré les conséquences de cette décision et estimé que le juge judiciaire avait l'obligation de garantir à la personne placée dans des conditions indignes de détention un recours préventif et effectif permettant de mettre un terme à la violation de l'article 3 de la Convention, en tant que gardien de la liberté individuelle, en application de l'article 66 de la Constitution. Cet arrêt de principe a ainsi ouvert une nouvelle voie de recours aux personnes détenues sans que le législateur ait eu l'occasion d'intervenir.

qu'il incombait « au législateur de garantir aux personnes placées en détention la possibilité de saisir le juge de conditions de détention contraires à la dignité de la personne humaine, afin qu'il y soit mis fin », ce que les procédures actuelles de référé ne permettaient pas. Il a en conséquence décidé l'abrogation, à compter du 1 mars dernier, du second alinéa de l'article 144-1 du code de procédure pénale en ce qu'il ne prévoyait pas un tel recours. Le Sénat a, à plusieurs reprises, interrogé le Gouvernement sur les suites qu'il entendait donner à cette décision et sur le dispositif qu'il envisageait de soumettre au législateur. Je dois à cet égard souligner combien notre collègue Jean-Pierre Sueur s'est investi sur le sujet, appelant plusieurs fois l'attention du Gouvernement. Les

Mais rendons à César ce qui lui appartient : ce texte est le fruit des réflexions de la Chancellerie sur le sujet, dont j'ai partagé l'analyse. Le dispositif envisagé me semble répondre en tous points aux demandes tant de la Cour européenne des droits de l'homme que du Conseil constitutionnel. Selon l'article unique du texte, toute personne détenue se plaignant de conditions indignes de détention aura le choix de saisir soit le juge administratif des référés, qui dispose d'un pouvoir d'injonction, soit le juge judiciaire, qui n'a pas un tel pouvoir mais qui peut éventuellement ordonner une remise en liberté. Concernant les critères de recevabilité de la demande, les allégations figurant dans la requête devront être circonstanciées, personnelles et actuelles. Le juge fera procéder aux vérifications nécessaires et recueillera les observations de l'administration pénitentiaire dans un délai compris entre trois et dix jours ouvrables. Si le juge estime la requête fondée, il reviendra d'abord à l'administration pénitentiaire de prendre des mesures pour mettre fin aux conditions de détention indignes. Le juge fera connaître à l'administration pénitentiaire les conditions de détention qu'il estime indignes, puis il lui fixera un délai, compris entre dix jours et un mois, pour y mettre fin par les moyens qu'elle estimera appropriés. L'administration pénitentiaire pourra notamment décider le transfèrement du détenu, avec l'accord du magistrat chargé du dossier s'il s'agit d'un prévenu. C'est seulement si le problème n'a pas été résolu par l'administration pénitentiaire dans le délai prescrit que le juge judiciaire sera alors amené à statuer pour mettre fin à ces conditions de détention. Il aura le choix entre trois options : ordonner le transfèrement de la personne détenue ; ordonner la mise en liberté de la personne placée en détention provisoire, éventuellement assortie d'un contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence sous surveillance électronique (ARSE) ; ordonner un aménagement de peine si la personne est éligible à une telle mesure. Toutefois, le juge pourra refuser de prendre l'une de ces trois décisions si le détenu a au préalable refusé un transfèrement proposé par l'administration pénitentiaire, sauf s'il s'agit d'un condamné et que ce transfèrement porterait une atteinte excessive à sa vie privée et familiale. La décision du juge pourra faire l'objet d'un appel, selon les cas devant la chambre de l'instruction ou devant la chambre de l'application des peines. L'appel du ministère public lui-même sera suspensif lorsqu'il sera formé dans un délai de vingt-quatre heures, l'affaire devant être examinée au plus tard dans un délai de quinze jours. Nous proposons qu'un décret en Conseil d'État vienne préciser les modalités de saisine du juge des libertés et de la détention (JLD) ou du juge de l'application des peines (JAP), ainsi que la nature des vérifications que le juge pourrait ordonner et l'articulation entre l'intervention du juge judiciaire et celle du juge administratif. administratif. Certains pourront regretter les conditions d'urgence de cet examen parlementaire, mais elles s'expliquent à la fois par la nécessité de ne pas laisser perdurer une carence législative trop longtemps, alors même que l'abrogation décidée par le Conseil constitutionnel est entrée en vigueur la semaine dernière,

Elle introduit dans notre code de procédure pénale une nouvelle voie de recours garantissant à chaque détenu la possibilité de faire constater des conditions indignes de détention afin qu'il y soit mis fin. Elle mettra notre législation en conformité avec la décision du Conseil constitutionnel du 2 octobre dernier, qui nous a donné jusqu'au 1 mars 2021 pour créer cette nouvelle voie de recours. Le Sénat est depuis longtemps attentif au problème de la condition carcérale. Je ne remonterai pas jusqu'aux discours de notre illustre prédécesseur Victor Hugo, qui, tout au long de sa carrière, a dénoncé l'inhumanité des des prisons du XIX siècle. Je préfère vous renvoyer sur ce point à l'excellent ouvrage de notre non moins excellent collègue Jean-Pierre Sueur, publié en 2018. Plus près de nous, comment ne pas évoquer le rapport rédigé en l'an 2000 par nos anciens collègues Jean-Jacques Hyest et Guy-Pierre Cabanel, qui avait contribué à la prise de conscience par les pouvoirs publics et par nos concitoyens de l'état si dégradé de notre parc pénitentiaire ? Depuis lors, des progrès ont été réalisés, grâce à des programmes successifs de rénovation et de construction de nouvelles places de prison. Depuis trois ans est mis en oeuvre le programme « 15 000 », qui doit aboutir à l'ouverture de 7 000 places d'ici à 2022 de 8 000 places supplémentaires à l'horizon de 2027. En outre, l'administration pénitentiaire a bénéficié de recrutements, notamment pour réduire le nombre de vacances de postes parmi les surveillants. Pourtant, des problèmes importants demeurent, notamment dans les maisons d'arrêt, qui restent suroccupées. Quand on regarde les chiffres, on peut avoir l'illusion que la situation s'est améliorée depuis un an. Le taux d'occupation de nos établissements pénitentiaires s'établit aujourd'hui à 105 %, alors qu'il était de 115 % au début de l'année 2020, et le nombre de matelas au sol, qui est de l'ordre de 740, a baissé de 60 % en un an. Il convient cependant de ne pas se tromper dans l'interprétation de ces chiffres. Ceux-ci s'expliquent en grande partie par la crise sanitaire, qui a entraîné la libération anticipée de nombreux détenus et qui a réduit les entrées en détention du fait du fonctionnement ralenti des juridictions pénales. Depuis plusieurs mois, on observe une remontée du nombre de détenus, qui est la conséquence logique de la reprise de l'activité dans nos juridictions. Il est à craindre que la surpopulation carcérale ne redevienne rapidement d'actualité. J'ajoute que la situation est particulièrement préoccupante dans plusieurs de nos établissements pénitentiaires d'outre-mer. Lors d'un déplacement en 2019, une délégation de la commission des lois avait par exemple pu constater les problèmes de surpopulation, d'hygiène et de violence dans l'établissement pénitentiaire de Guyane. Je ne doute pas que nous aurons l'occasion d'y revenir au cours de la discussion. Les peines d'emprisonnement privent les individus de leur liberté, mais elles ne doivent pas les dépouiller de leur dignité. Pour notre pays, il s'agit d'un enjeu non seulement de respect des droits fondamentaux, mais aussi de sécurité, puisque l'on ne peut pas travailler efficacement à la réinsertion des détenus et lutter contre la récidive si les conditions de détention sont inacceptables. La proposition de loi qui vous est soumise ouvre une nouvelle voie de recours, organisée en trois grandes étapes. D'abord, le détenu dépose une requête, examinée soit par le juge des libertés et de la détention si la personne est placée en détention provisoire, soit par le juge de l'application des peines s'il s'agit d'un condamné. Le juge fait procéder aux vérifications nécessaires et il recueille les observations de l'administration pénitentiaire. Ensuite, s'il estime la requête fondée, le juge fait connaître à l'administration pénitentiaire les conditions de détention qu'il considère indignes et il lui fixe un délai pour y mettre fin. C'est donc dans un premier temps l'administration pénitentiaire qui doit faire le nécessaire pour remédier au problème. Il lui revient de déterminer les moyens à mettre en oeuvre, le juge judiciaire ne pouvant pas lui adresser d'injonction, ce qui est conforme à la répartition des compétences habituelle entre les deux ordres de juridiction. de juridiction. Enfin, si l'administration pénitentiaire ne parvient pas à résoudre le problème dans le délai imparti, le juge prend une décision pour mettre un terme aux conditions indignes de détention. Il a la possibilité d'ordonner le transfèrement de la personne détenue, d'ordonner sa remise en liberté s'il s'agit d'une personne placée en détention provisoire ou d'ordonner un aménagement de peine si la personne est définitivement condamnée, à condition qu'elle soit éligible à une telle mesure. Toutefois, le juge peut refuser de prendre l'une de ces trois décisions si le détenu a, au préalable, refusé un transfèrement proposé par l'administration pénitentiaire, sauf s'il s'agit d'un condamné et que ce transfèrement aurait porté une atteinte excessive à sa vie privée et familiale. En d'autres termes, le juge peut décider qu'un détenu qui aura refusé sans motif valable la solution d'un transfèrement restera en détention. Vous le voyez, mes chers collègues, la proposition de loi ne consacre pas un droit absolu à la remise en liberté. Elle cherche à concilier le droit à des conditions dignes de détention avec le droit à la sûreté et avec l'objectif de prévenir les atteintes à l'ordre public. Dans le texte qu'elle a élaboré, la commission des lois s'est attachée à préciser les hypothèses dans lesquelles il est possible de former un recours en appel. Il est notamment important que le détenu puisse contester la décision du juge de déclarer son recours irrecevable, ce qui n'était pas prévu dans le texte initial. Je précise que l'appel est examiné, selon les cas, par le président de la chambre de l'instruction ou par le président de la chambre de l'application des peines. Sur mon initiative, la commission a également souhaité mieux associer le juge d'instruction à la procédure, en prévoyant d'abord qu'il soit informé du dépôt de la requête, puis qu'il puisse être consulté par le JLD avant de rendre sa décision. Le juge d'instruction peut en effet avoir connaissance d'informations utiles pour éclairer l'appréciation qu'il convient de porter sur le dossier. La proposition de loi déposée par François-Noël Buffet cosignée par des collègues membres des groupes Les Républicains, Union Centriste, Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, Rassemblement Démocratique et Social Européen, Les Indépendants - République et Territoires, Écologiste - Solidarité et Territoires. Cela montre qu'elle bénéficie d'un large soutien. Par la voix de notre collègue Jean-Pierre Sueur, le groupe socialiste a regretté que nous n'ayons pas pris le temps de rédiger un texte de consensus qui aurait pu recevoir un soutien encore plus large. Je comprends l'intérêt qu'aurait pu présenter une telle démarche : elle aurait donné une force encore plus grande au texte issu des délibérations du Sénat. Je note cependant qu'elle aurait ralenti le rythme de nos travaux, alors que l'échéance du 1 mars, fixée par le Conseil constitutionnel, est déjà dépassée. J'observe surtout- le débat au sein de notre commission le 3 mars l'a bien montré -qu'il existe un accord entre nous sur les grands principes, mais que des divergences, tout à fait légitimes au demeurant, subsistent sur les modalités pratiques de la réforme. concernant les critères de recevabilité de la requête, le texte demande que celle-ci contienne des allégations circonstanciées, personnelles et actuelles, constituant un commencement de preuve. favorable à un assouplissement de ces critères, monsieur Sueur, ce qui pourrait poser à mon avis un problème au regard du principe de bonne administration de la justice, avec le risque que les magistrats ne soient submergés par des demandes peu étayées, uniquement motivées par le souci de faire libérer un détenu par le biais de cette nouvelle voie de recours. Une deuxième divergence demeure sur la place à accorder au transfèrement. Le transfèrement nous paraît préférable à une libération, qui doit rester la solution de dernier ressort, et il peut constituer une solution appropriée si un établissement est saturé mais que d'autres établissements à proximité sont moins chargés. Or vous défendez des propositions qui ont pour objectif commun de rendre plus difficile le transfèrement en multipliant les conditions à satisfaire. Il s'agit là- nous y reviendrons sans doute -d'une vraie différence d'appréciation entre nous. Pour terminer, je tiens à remercier François-Noël Buffet d'avoir pris l'initiative de déposer cette proposition de loi. Je salue la décision du Gouvernement d'avoir inscrit ce texte à l'ordre du jour de nos deux assemblées en vue de son adoption rapide. J'invite l'ensemble de nos collègues à l'approuver, afin de remédier à la lacune qui a été identifiée dans la garantie de nos droits fondamentaux. Je forme le voeu que ce texte marque une nouvelle étape sur la voie d'un redressement durable de notre service public pénitentiaire, l'objectif essentiel étant d'améliorer concrètement les conditions de détention, avec l'espoir que cette amélioration rende un jour à peu près inutile la nouvelle voie de recours dont nous débattons aujourd'hui. La parole

monsieur le président de la commission des lois, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, il est une certitude qui m'a accompagné durant toute ma vie d'avocat conduit, désormais garde des sceaux, à agir : la privation de liberté ne doit pas être, ne peut pas être, une privation de dignité. Car nier les droits fondamentaux des personnes revient à contester leur humanité même ! Plus elle désocialise et déshumanise, plus la prison est un vecteur de récidive. La peine doit évidemment avoir un sens. C'est bien tout l'objet de mon action depuis mon arrivée à la tête du ministère de la justice. J'ai d'abord souhaité que l'on poursuive activement l'accompagnement des dispositions de la loi du 23 mars 2019, qui a refondé l'échelle des peines, en en restreignant la possibilité de prononcer des emprisonnements de courte durée, qui n'ont que pour effet la désocialisation, et en favorisant le recours aux alternatives à l'incarcération pour les actes les moins graves. Vous le savez, la crise sanitaire a entraîné une réduction inédite de la population carcérale. Mais, depuis la reprise de l'activité juridictionnelle, le nombre de détenus augmente à nouveau. Nous comptabilisons 5 000 détenus de plus depuis le premier déconfinement, et 849 détenus sont aujourd'hui contraints de dormir sur des matelas posés à même le sol. Nous devons mettre un terme à cette situation par une politique carcérale cohérente et volontariste. Nous ne pouvons pas perdre cette possibilité d'une population pénale maîtrisée offrant à la fois de meilleures conditions de détention comme de travail pour les personnels pénitentiaires. J'ai donc réuni très récemment l'ensemble des chefs de cour et de juridiction pour qu'ils analysent attentivement les marges de progression et qu'ils adaptent rapidement la politique pénale dans chacun de leur ressort. Les aménagements de peine dès leur prononcé ont très significativement augmenté, de 3 % à 11 % en moins d'un an. C'est un signe très positif dont nous devons collectivement nous réjouir. Cependant, il convient de redoubler d'efforts. La loi du 23 mars et de réforme pour la justice porte en elle une révolution, certes juridique, mais aussi et peut-être surtout culturelle. Elle implique que l'ensemble des acteurs de la chaîne pénale- autorité judiciaire, services pénitentiaires, mais aussi avocats -adaptent leurs pratiques. Le travail engagé doit se poursuivre quand on songe que, depuis l'entrée en vigueur du « bloc peine », au mois de mars 2020, qui interdit les peines de prison de moins d'un mois, 227 peines illégales ont tout de même été prononcées. J'ai par ailleurs souhaité que les alternatives à la détention soient développées en amont, c'est-à-dire au stade de l'opportunité des poursuites, car il ne faut pas confondre toutes les délinquances. La réponse pénale doit ainsi être adaptée, et la prison en fait évidemment partie, lorsqu'il s'agit de délinquance organisée et de violences graves aux personnes. Mais elle doit également prendre en compte la délinquance du quotidien, dite de « basse intensité », mais qui pourrit la vie de nos concitoyens. Cette dernière doit d'abord être traitée avec célérité et efficacité pour garantir la pédagogie de la réponse pénale, qui doit permettre de rompre le cercle vicieux de la délinquance. La prison neutralise, mais, souvent, elle désocialise. Elle est parfois criminogène. Pour les incivilités et les délits de faible gravité, il faut des réponses rapides et constructives. C'est tout l'objet de la politique de justice de proximité que je porte et à laquelle la proposition de loi du même nom que j'ai défendue devant vous a fait écho. L'amélioration des conditions de détention passe également par la construction de nouvelles places de prison pour écrouer dans des conditions plus dignes. Nous allons construire 15 000 places supplémentaires, conformément aux engagements du Président de la République. Les 7 000 premières places du programme immobilier pénitentiaire sont résolument engagées. L'objectif est désormais de lancer les 8 000 places supplémentaires avant le terme de la mandature, avec une livraison prévue à l'horizon de 2027. J'annoncerai d'ailleurs dans les jours à venir les sites qui ont été retenus par mes services. Il nous faut enfin, et c'est l'objet de ma présence devant vous cet après-midi, tirer toutes les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel du 2 octobre 2020, qui demandait au législateur de garantir aux détenus placés en détention provisoire la possibilité de saisir le juge de conditions de de détention indignes. Cette décision fait suite à un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 30 janvier 2020 ayant condamné la France pour ses conditions de détention dans plusieurs établissements pénitentiaires, ainsi qu'à deux arrêts de la Cour de cassation du 8 juillet 2020. Afin de mettre notre droit en conformité avec les exigences constitutionnelles, j'ai immédiatement mobilisé mes services pour concevoir ce recours effectif. Conscient des enjeux, j'ai souhaité le soumettre à l'avis du Conseil d'État dès le 1 décembre 2020. L'amendement reprenant ce dispositif ainsi validé par le Conseil d'État a été déposé à l'Assemblée nationale lors de l'examen du projet de loi relatif au Parquet européen au mois de décembre dernier. Pour faciliter les débats, je l'avais transmis en parallèle aux commissions des lois du Sénat et de l'Assemblée

cet amendement a été déclaré irrecevable. Depuis lors, le Conseil constitutionnel a une nouvelle fois été saisi sur les conditions de détention par une nouvelle QPC, actuellement pendante devant lui, concernant cette fois les détenus condamnés. Je le dis d'emblée, il nous faudra peut-être adapter notre réponse même si nous avions anticipé cette situation en prévoyant un recours effectif tant pour les prévenus que pour les condamnés incarcérés. Tel est donc l'objet de la proposition de loi que vous examinez ; elle enrichit le dispositif que nous avions conçu.

ainsi qu'à l'article 707 pour les condamnés. Si la personne est en détention provisoire, la juridiction compétente pour statuer sur la demande sera le juge des libertés et de la détention. Si la personne est en exécution de peine, la requête relèvera alors de la compétence du juge de l'application des peines. Le juge saisi pourra, si nécessaire, faire vérifier les allégations circonstanciées du détenu, le texte reprenant les formulations des arrêts de la Cour de cassation ; s'il estime la requête justifiée, il fixera le délai dans lequel l'administration pénitentiaire devra mettre fin aux conditions indignes de détention, le cas échéant en transférant la personne dans un autre établissement pénitentiaire. Si les conditions indignes perdurent à l'issue de ce délai, le juge pourra ordonner lui-même un transfèrement ou, pour les prévenus, la libération de la personne, le cas échéant sous mesure de sûreté. Pour les condamnés, il pourra prononcer une libération sous aménagement de peine, si la personne est éligible à une telle mesure. Le texte prévoit toutefois que la personne ne pourra pas être libérée si elle s'oppose au transfèrement qui lui aura été proposé, sous réserve, pour les condamnés, de la nécessité de ne pas porter une atteinte excessive au droit au respect de sa vie familiale. Ce nouveau dispositif répond ainsi aux exigences constitutionnelles et permet de trouver un équilibre pour que le service public de la justice continue de fonctionner, en assurant la sécurité de tous. La situation de nos prisons nous oblige collectivement à porter cette exigence d'humanité et d'efficacité pour maintenir la justice au coeur de notre pacte républicain.

la privation de liberté ne doit en aucun cas remettre en cause la dignité de l'être humain.

qu'est-ce qui vous a empêché, entre le 2 octobre et le 1 mars, de déposer un projet de loi ? Je l'ai dit ! Rien !

Il semble au contraire avoir pour objectif principal »- j'insiste sur cette expression -« de limiter les conséquences des jurisprudences, en faisant obstacle aux recours qu'elles créent et même en restreignant les prérogatives du juge au profit de celles de l'administration. Je vais citer cinq points évoqués dans cette lettre ; ils sont repris par l'Observatoire international des prisons et de nombreux magistrats et avocats que nous avons reçus,

l'arrêt qui, en présence d'une description circonstanciée, s'arrête au fait qu'elle ne renverrait qu'aux conditions générales de détention dans l'établissement pénitentiaire en cause et qui exige de l'intéressé qu'il démontre le caractère indigne de ses conditions personnelles de détention.

point -, les mesures appropriées pour améliorer les conditions de détention échappent en grande partie au contrôle du juge,

combiné à la surpopulation carcérale qui touche de nombreux établissements, ne manquera pas de conduire au placement d'une autre personne dans les conditions contestées par le détenu transféré ; ce risque doit être expressément écarté par la loi. » loi. » Nous le savons, vous l'avez dit, et tout le monde le dit, il faut que la France applique ce que disent la Cour européenne des droits de l'homme et la Cour de cassation.

Or, à cet égard, il y a quelque chose de quand même très étonnant : à la suite de l'ordonnance du 25 mars 2020, plus de 13 000 détenus ont été libérés, et nous sommes redescendus en

la proposition de loi du président Buffet que nous examinons cet après-midi tire les conséquences d'une récente décision du Conseil constitutionnel, qui a estimé qu'il incombait au législateur de garantir aux personnes placées en détention la possibilité de saisir le juge de conditions de détention contraires à la dignité de la personne, afin qu'il y soit mis fin. Cette décision du Conseil constitutionnel fait suite à un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme condamnant la France, ainsi qu'à un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation qui a créé une nouvelle voie de recours ouverte aux personnes placées en détention provisoire. La proposition de loi reprend le dispositif d'un amendement que le Gouvernement avait initialement envisagé de faire adopter, en décembre 2020, par l'Assemblée nationale dans le cadre de l'examen du projet de loi relatif au Parquet européen. Le Gouvernement a cependant dû y renoncer, lorsque l'amendement a été déclaré irrecevable par l'Assemblée nationale sur le fondement de l'article 45 de la Constitution. Toujours est-il que la décision du Conseil constitutionnel imposait une action rapide, dans le délai qu'il avait prescrit. C'est ce qui a conduit notre collègue François-Noël Buffet à prendre l'excellente initiative du dépôt de cette proposition de loi. Le texte insère dans le code de procédure pénale un nouvel article 803-8, qui prévoit dans quelles conditions et selon quelles modalités un détenu peut saisir le juge judiciaire, lorsqu'il estime subir des conditions indignes de détention, afin qu'il y soit mis fin. Il procède également à une mesure de coordination à l'article 144-1 du code de procédure pénale et complète le paragraphe III de l'article 707 du même code. Ce paragraphe III affirme le droit, pour toute personne condamnée incarcérée en exécution d'une peine privative de liberté, de bénéficier, chaque fois que cela est possible, d'un retour progressif à la liberté, en tenant compte des conditions matérielles de détention et du taux d'occupation de l'établissement pénitentiaire, dans le cadre d'une mesure de semi-liberté, de placement à l'extérieur, de détention à domicile sous surveillance électronique, de libération conditionnelle ou d'une libération sous contrainte, afin d'éviter une remise en liberté sans aucune forme de suivi judiciaire. La proposition de loi précise que le droit de la personne d'être incarcérée dans des conditions respectant sa dignité est garanti par les dispositions du nouvel article 803-8. Je me réjouis que la commission ait approuvé le dispositif équilibré de ce texte, tout en y apportant plusieurs précisions pour le parfaire.

l'adoption de cette proposition de loi ne résoudra pas à elle seule le problème posé par les conditions de détention dans notre pays. Elle ne dispensera donc pas la France de poursuivre son programme de construction et de rénovation de places de prison- vous en avez parlé, monsieur le Je veux ici rappeler que le Gouvernement s'est engagé à ouvrir 7 000 places d'ici à 2022 et à lancer les opérations pour l'ouverture de 8 000 places supplémentaires à l'horizon de 2027. À plusieurs reprises, dans le cadre des travaux de la commission des lois, notamment en tant que rapporteur pour avis du budget de l'administration pénitentiaire, j'ai eu l'occasion de m'interroger sur le manque d'ambition de ce programme, qui se contente de prolonger des projets lancés par la précédente majorité.

Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, cela fait des années que nous ne cessons de décrier le sort réservé aux détenus dans les prisons françaises. Entre surpopulation carcérale et conditions de détention inhumaines et dégradantes, nos prisons ne sont plus, depuis bien trop longtemps maintenant, à l'image d'un pays qui se revendique patrie des droits de l'homme ... et de la femme- nous sommes le 8 mars, Les chiffres sont alarmants : en moins de vingt ans, les prisons françaises sont passées de 48 000 à 72 000 personnes détenues. Si ce chiffre a récemment connu une légère baisse liée à la crise sanitaire, il n'en reste pas moins qu'au 1 janvier 2021 ce sont plus de 20 000 personnes qui sont encore détenues dans des établissements, dont le taux d'occupation est supérieur à 120 %. En outre, à ce jour, une trentaine d'établissements pénitentiaires a été considérée par la justice comme exposant les personnes détenues à des traitements humiliants. Cette situation, nous ne pouvons pas prétendre la découvrir aujourd'hui Déjà en 2018, j'interpellais le Gouvernement sur les violences et les mauvais traitements que subissaient certains détenus à la prison de Villefranche-sur-Saône. La garde des sceaux d'alors m'avait formulé une réponse qui était le symbole du déni ordinaire des pouvoirs publics face à ce sujet pourtant si important, mais peu traité par les médias, donc peu exposé au regard des citoyens. En juillet 2019, je publiais une tribune dans la presse pour dénoncer les graves violences physiques et morales qui ont lieu dans nos prisons et, à de nombreuses autres occasions, nous avons publiquement défendu le droit au respect de la dignité en prison, y compris dans cet hémicycle. Ces nombreux appels sont restés lettre morte jusqu'aux décisions de la CEDH du 30 janvier 2020 et surtout du Conseil constitutionnel du 2 octobre dernier- c'est à cette dernière décision que nous devons ce texte précipitamment mis à l'ordre du jour de notre chambre. a considéré qu'il incombait au législateur de garantir aux personnes placées en détention la possibilité de saisir le juge pour des conditions de détention contraires à la dignité de la personne humaine. L'échéance avait été fixée au 1 mars 2021. Parce que la défense de la dignité des personnes détenues est notre engagement de longue date, nous ne pouvons que soutenir cette proposition de loi et nous y associer. N'oublions pas que, derrière celle-ci, des vies sont concernées. La récente actualité nous le rappelle clairement. Le 2 février dernier, un homme incarcéré à Meaux est décédé il avait été hospitalisé quelques jours plus tôt à la suite d'une violente altercation avec des surveillants. Le même jour, à la maison d'arrêt pour femmes de Poitiers-Vivonne, une violente altercation avec des surveillantes causa à une détenue quarante-deux jours d'ITT. Monsieur le garde des sceaux, selon votre prédécesseure, l'objectif du Gouvernement était, je cite, que, « d'ici à la fin du quinquennat, des conditions de détention plus dignes et conformes aux engagements européens soient mises en place ». de loi est une première étape, nous attendons toutefois une amélioration urgente des conditions de vie dans les lieux de détention, ainsi que des relations entre les personnes détenues et les surveillants. Nous attendons aussi davantage d'écoute de la part du personnel médical et d'encadrement de ces

Ce n'est pas en construisant de nouvelles prisons, sitôt construites, sitôt remplies, que l'on réglera le problème de la surpopulation carcérale.

c'est un constat que nous avons tous fait cet après-midi : la France fait partie des États européens dont les prisons sont les plus encombrées et dont la population pénale augmente. Au 1 janvier 2020, elle comptait 70 651 détenus pour 61 080 places opérationnelles, portant ainsi la densité carcérale globale à 115,7 %. Alors Alors même que le principe d'encellulement individuel est inscrit dans notre droit depuis 1875, cette surpopulation chronique emporte de graves conséquences sur les droits et la dignité des détenus. Entre 2015 et 2017, trente-deux requêtes ont été déposées par des personnes détenues en métropole et en outre-mer auprès de la Cour européenne des droits de l'homme, laquelle a, le 30 janvier 2020, condamné notre pays à résorber l'inflation carcérale et à instituer un recours préventif et effectif, permettant aux personnes détenues de faire cesser ces atteintes graves à leurs droits fondamentaux. Dans un arrêt du 8 juillet 2020, la Cour de cassation, concernant un placement en détention provisoire, posait le principe selon lequel des conditions indignes de détention sont susceptibles de constituer un obstacle à la poursuite de cette détention. Cette solution, entre maintien en détention et libération sèche, ne pouvait pas être considérée comme satisfaisante. Aussi, saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a, le 2 octobre dernier, décidé l'abrogation à la date du 1 mars 2021 du second alinéa de l'article 144-1 du code de procédure pénale, qui prévoyait la remise en liberté d'une personne placée en détention provisoire, lorsque les conditions de ce placement cessaient d'être remplies. Il laissait par conséquent six mois au législateur pour faire respecter ce droit à être incarcéré dans des conditions qui ne violent pas la dignité humaine. La présente proposition de loi, sur laquelle le Gouvernement a engagé la procédure accélérée, tire les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel, en créant un dispositif équilibré, à la fois protecteur des droits des détenus et garant de la sécurité des Français. S'inscrivant dans une démarche transpartisane initiée par le président Buffet, que je remercie, elle s'inspire de la proposition que vous aviez, monsieur le garde des sceaux, communiquée pour avis au Conseil d'État le 1 décembre dernier et dont la commission des lois avait été destinataire. Son adoption sous forme d'amendement à l'Assemblée nationale dans le cadre de l'examen du projet de loi relatif au Parquet européen n'a pas été possible, car cet amendement a été déclaré irrecevable au regard de l'article 45 de notre Constitution. Je ne pense pas qu'il soit utile de gloser sur le retard pris dans le vote de ces dispositions. Il me semble que la responsabilité est collective. Je crois utile de rappeler que l'initiative de la loi appartient également au Parlement. Cette parenthèse refermée, le dispositif créé ne constitue pas à lui seul la solution pour améliorer les conditions de détention dans notre pays- nous en sommes tous d'accord. Ces dernières années, des mesures ont été prises pour incarcérer plus dignement. S'il est vrai que l'incarcération est nécessaire dans certains cas, la peine est bien la privation de la liberté, et non la privation de la dignité, comme vous l'avez indiqué, monsieur le garde des sceaux. Le Président de la République s'est engagé à créer 15 000 places de prison d'ici à 2027 ; 7 000 sont en cours de livraison. Je salue d'ailleurs la création de 981 places de prison supplémentaires en outre-mer ces dernières années, dont 182 dans mon département. Un rapport de 2014, commandé par l'ancienne garde des sceaux, Mme Christiane Taubira, avait dressé un constat particulièrement alarmant sur le surpeuplement de certains établissements ultramarins. Ces constructions ont permis de réduire le taux moyen d'occupation carcérale dans ces territoires À l'horizon de 2026, nous attendons 1 156 places supplémentaires. Néanmoins, la prison n'est pas la seule solution, et je me félicite que des alternatives à la détention soient aussi développées. C'est le sens d'une réponse pénale adaptée, proposée chaque fois qu'elle est possible et utile. Le groupe RDPI votera donc en faveur de cette proposition de loi, qu'il a cosignée et qui permet un recours effectif devant le juge judiciaire pour faire constater des conditions de détention contraires à la dignité humaine et y mettre fin. Il est bien évident que les mesures mises en place pour désengorger les prisons doivent être poursuivies.

Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, dès 2013, la France a été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme en raison des conditions de détention d'un détenu qui, à la différence de nombreux autres demeurés silencieux, avait porté sa réclamation jusqu'à l'une des instances internationales les plus influentes. Permettez-moi de rappeler quelques éléments qui furent relevés à l'occasion de cette décision au sujet des conditions de détention

le local des douches était insalubre avec seulement une petite fenêtre et aucun système d'aération ; des cafards couraient partout. Cette description est absolument édifiante, mais nous ne l'apprenons pas aujourd'hui. En plus d'un phénomène de surpopulation, le milieu carcéral est insalubre. En cette Journée internationale des droits des femmes, j'aurai également une pensée pour les nombreuses femmes détenues dans notre pays, qui subissent des conditions similaires. Évidemment, il n'est nullement question de remettre en cause le principe même de l'incarcération. Aux délits sont associées des peines, parmi lesquelles la prison. celle-ci ne peut pas avoir pour fonction d'humilier les détenus. Nous devons tous avoir à l'esprit que chacun a vocation à en sortir. Nous espérions que ce constat et cette condamnation, en 2013, permettent d'améliorer l'état de nos prisons. Tel n'a pas été le cas. plus de subir des conditions de détention indignes et de souffrir des conséquences de la surpopulation carcérale, les détenus ne disposent d'aucun moyen de les faire cesser. En raison de cela, la France a été condamnée une première fois par la CEDH en mai 2015. C'est également pour ce motif qu'elle l'a été une nouvelle fois en 2020. Dans cette dernière décision, les juges européens ont rappelé trois objectifs à l'État français : supprimer le surpeuplement dans les établissements pénitentiaires ; améliorer les conditions de détention ; établir un recours effectif. Ce tableau, que je viens brièvement de dépeindre, n'est pas à l'honneur de notre nation. Aussi, il y a lieu de se réjouir de l'initiative du Sénat qui vise à y mettre fin.

Un droit de recours effectif ne répare pas des canalisations bouchées, pas plus qu'il ne désinsectise une cellule ou qu'il ne permet d'aérer des douches collectives. Déplacer les détenus d'une maison d'arrêt à une autre, comme par un jeu de chaises musicales, ne permet pas non plus de réduire le nombre de détenus par maison d'arrêt. Tout cela est et demeurera une question de moyens matériels, bien au-delà des moyens juridictionnels. Renforcer les droits des prisonniers est une chose ; s'assurer que leur place est réellement en prison en est une autre. Le Sénat y travaille aussi, et nous aurons d'ailleurs demain

cette proposition de loi arrive tardivement, mais elle a au moins le mérite d'arriver, après une série de décisions d'instances européennes et nationales relevant de graves atteintes aux droits et à la dignité des personnes détenues. La condamnation historique de la France, le 30 janvier 2020, par la Cour européenne des droits de l'homme a conduit à l'indemnisation de trente-deux personnes incarcérées dans différents centres pénitentiaires, en métropole et outre-mer,

nécessitaient des mesures de réorganisation du service public de la justice. Cette décision forte a eu pour conséquence un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation, qui a estimé, le 8 juillet 2020, que le juge judiciaire avait l'obligation de garantir à la personne placée dans des conditions indignes de détention un recours préventif et effectif, sans que le législateur intervienne. Cette situation a été jugée insatisfaisante par le Conseil constitutionnel, qui a donc affirmé, en octobre dernier, qu'il incombait au législateur de garantir aux personnes placées en détention la possibilité de saisir le juge de conditions de détention contraires à la dignité de la personne humaine afin qu'il y soit mis fin. la présente proposition de loi tire les conséquences de cette censure et prévoit un dispositif de nature à garantir le droit à des conditions dignes de détention.

Malgré le caractère extrêmement grave des causes qui ont conduit à légiférer, bien tardivement, et même si je peux partager, pour une bonne partie, les propos de Jean-Pierre Sueur, je tiens à exprimer notre satisfaction de voir aujourd'hui cette question abordée avec des mesures générales pour mettre fin à cette situation inacceptable. C'est pourquoi nous voterons en faveur de cette proposition de loi. Néanmoins, il est primordial de rappeler que le profond décalage entre les normes applicables et la réalité quotidienne des conditions de vie des personnes détenues n'a que trop duré, comme le notait le Contrôleur général des lieux de privation rapport en 2018 : « Ni les lois sur l'encellulement individuel ni les normes relatives à l'espace vital par personne détenue, telles que recommandées par le Comité européen de prévention de la torture, ne sont respectées, pas plus que ne le sont les propres normes de l'administration pénitentiaire. » » Permettez-moi enfin, monsieur le garde des sceaux, de condamner, en cette Journée internationale des droits des femmes, les mauvaises conditions de vie des femmes en prison, qui portent trop souvent atteinte à leur dignité. La construction de nouvelles places de prison, comme le souligne le président de la commission des lois, auteur de la proposition de loi, à la fin de l'exposé des motifs, ne peut être une réponse satisfaisante au problème. C'est pourtant, hélas, ce que vous proposez. Vous souhaitez également mettre fin aux réductions automatiques de peines en les assortissant de conditions, relative à la bonne conduite existant déjà. Or, comme le signalait hier la Contrôleuse générale des lieux de privation de liberté, Dominique Simonnot : « Il y a sans doute beaucoup de détenus qui voudraient être soignés, trouver un boulot ou une formation en prison, ... Bien sûr ! ... mais on ne leur en donne pas les moyens. » de prendre des mesures qui ne feront qu'aggraver les conditions de détention, il est au contraire urgent, selon nous, de réfléchir globalement au système pénal que nous souhaitons pour notre pays. pays. Les études sur le sujet sont unanimes : la seule manière de lutter contre la surpopulation carcérale, et donc contre les conditions de détention indignes, est d'engager un grand plan de décroissance carcérale. Cela irait à rebours des choix des gouvernements successifs, prôné une plus grande sévérité en matière de répression et une plus grande rapidité dans l'exécution des réponses pénales : alourdissement des peines et de la fermeté des sanctions prononcées par les juridictions, d'un côté ; extension du champ d'action de la procédure de comparution immédiate et volonté de mise à exécution des peines, de l'autre. Il faut y ajouter l'augmentation du nombre de personnes placées en détention provisoire. Seule la mise en place d'une politique publique de désinflation carcérale sera en mesure de mettre un terme aux échecs des politiques antérieures. Cette proposition de loi doit entrer en vigueur rapidement, mais, surtout, ouvrir la voie à un débat plus large en la matière et à

collègue François-Noël Buffet, qui vise à faire cesser une situation insupportable pour le pays des droits de l'homme. Prenant acte des divers arrêts et sanctions visant notre République, cette proposition a deux objets principaux. Le premier, c'est de garantir à tous les détenus des conditions de détention compatibles avec le principe de dignité de la personne humaine. Le second, c'est de créer une voie de recours effective lorsque sa dignité est bafouée.

Depuis le début des années 2000, le nombre de détenus en France a augmenté chaque année, alors que, pendant cette période, le nombre de places supplémentaires a crû moins vite, voire a diminué dans certains établissements. Quand, en Allemagne ou au Royaume-Uni, la population carcérale des établissements pénitentiaires demeure légèrement en deçà du taux d'occupation maximal, aux alentours de 96 % du nombre de places opérationnelles, nous sommes à 116

un rapport du Sénat, rédigé par nos anciens collègues Guy-Pierre Cabanel et Jean-Jacques Hyest évoquait « des prisons républicaines aux oubliettes de la société », « une honte et une humiliation pour la République ». En 2019, un rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté établissait que la densité moyenne des maisons d'arrêt en France était de 138 personnes pour 100 places opérationnelles, 44 de ces établissements ayant une densité supérieure à 150 %. Pour certains, le taux d'occupation peut aller jusqu'à 200 %, voire 213 %. Je pense ici au quartier de la maison d'arrêt du centre pénitentiaire de Ducos en Martinique. Cette situation est bien connue des pouvoirs publics depuis une dizaine d'années. Elle fait peser au-dessus de nos têtes une permanente épée de Damoclès. La France avait déjà été condamnée pour la première fois à ce sujet en 2013. Il s'agissait alors de la maison d'arrêt Charles-III de Nancy. Pour autant, nos établissements pénitentiaires sont toujours surpeuplés et, bien souvent, les conditions de détention au sein des maisons d'arrêt sont considérées comme indignes. Il est question de vétusté, d'insalubrité, de trop grande promiscuité. C'est En effet, alors que tout propriétaire privé doit légalement garantir à ses locataires une surface habitable d'au moins neuf mètres carrés, il n'est pas rare que l'État français fasse cohabiter plusieurs codétenus dans une cellule de huit mètres carrés, avec un ou plusieurs matelas au sol. Cette situation est indigne. Alors qu'en pleine crise sanitaire, pour assurer la protection de la santé de l'ensemble de nos concitoyens, des mesures drastiques de distanciation physique s'imposent à tous, depuis maintenant presque un an, l'opinion publique a découvert qu'il n'était pas rare que trois codétenus partagent la même cellule. C'est cette situation que vivaient bon nombre des trente-deux requérants qui ont intenté une action contre la France devant la Cour européenne des droits de l'homme.

ou traitements inhumains ou dégradants ». Pour le moment, nous échappons à la mise en oeuvre de la procédure dite de « l'arrêt pilote », une procédure qui permet d'identifier des problèmes structurels et, surtout,

de surpopulation carcérale, et je m'adresse ici au Gouvernement, la situation exige, comme le précise la Cour de Strasbourg, « l'adoption de mesures générales et structurelles visant à supprimer le surpeuplement et à améliorer les conditions matérielles de détention À la problématique des conditions de détention indignes, conséquence d'une surpopulation carcérale, s'ajoute la question du droit de recours effectif. Lorsque l'on a le sentiment que son droit à la dignité est bafoué, il n'y a rien de plus dramatique que le sentiment d'être abandonné par la Nation. En se mettant au diapason de la juridiction européenne, le Conseil constitutionnel, dans une décision qui brille par sa clarté et sa fermeté, est venu sanctionner le silence de la loi, le 2 octobre dernier. En avec la Cour de Strasbourg, qui a constaté, à raison, que le pouvoir d'injonction du juge des référés n'était que de portée limitée, notre juge constitutionnel a également sanctionné notre incompétence en considérant que, trop souvent, les recours dont disposent

En premier lieu, c'est à nous, législateurs, qu'il incombe de modifier la loi pour faire cesser cette anomalie. Ce sera, ensuite au Gouvernement, ou plus précisément à l'administration pénitentiaire, de prévenir au maximum toute atteinte à la dignité des personnes détenues. Enfin, il reviendra au juge judiciaire, garant de la liberté individuelle, de mettre en oeuvre toute mesure de nature à faire cesser une atteinte à la dignité lorsqu'il sera saisi d'une situation individuelle. Nous saluons encore une fois l'initiative prise par le président Buffet devant l'inaction du Gouvernement, alors que la date butoir fixée par le Conseil constitutionnel se rapprochait. Nous saluons également la qualité du travail réalisé par notre rapporteur, Christophe-André Frassa, qui a su, dans le temps très limité dont il disposait, proposer à notre commission des améliorations bienvenues. Vous l'aurez compris, mes chers collègues, en attendant que soit mise en oeuvre une réorganisation structurelle et profonde de notre service public pénitentiaire, le groupe Union Centriste soutiendra cette proposition de loi sans réserve. La parole

Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui intervient après l'arrêt de condamnation de la Cour européenne des droits de l'homme à l'encontre de la France du 30 janvier 2020. La France a alors été condamnée à indemniser trente-deux personnes incarcérées dans un certain nombre d'établissements pénitentiaires de métropole et d'outre-mer. La Cour européenne des droits de l'homme a notamment relevé des conditions indignes de détention de ces prisonniers, considérant

De même, elle a relevé la présence de nuisibles, tels que des cafards, des rats, des poux, des punaises ou autres parasites. Elle en appelle donc à traiter ces mauvaises conditions par des moyens plus appropriés de désinfection, des produits d'entretien, des fumigations et en procédant à des vérifications régulières des cellules, ainsi qu'à prendre des mesures visant à résorber véritablement la surpopulation carcérale. Cet arrêt de condamnation du 30 janvier 2020 relève enfin, et c'est là un point important, le non-respect de l'article 13 de la Convention européenne, qui reconnaît à toute personne dont les droits et libertés ont été violés un droit à un recours effectif devant une instance nationale. La Cour souligne en effet que les requérants ne disposent pas d'une voie de recours effective afin de faire cesser ces conditions de détention jugées indignes.

le Conseil constitutionnel a exigé du législateur qu'il garantisse aux personnes détenues la possibilité de saisir le juge de conditions de détention contraires à la dignité de la personne, et ce en votant une nouvelle loi avant le 1 mars 2021. S'il est évident que l'échéance ne sera pas respectée, la présente proposition de loi répond à un impératif de dignité humaine et constitue une étape importante pour améliorer le respect des droits fondamentaux dans notre pays.

monsieur le garde des sceaux, cette amélioration ne saurait faire perdre de vue ce qui doit être, me semble-t-il, la réponse véritable et durable à la question des conditions de détention, qui nous occupe aujourd'hui. Je veux parler de la construction de nouveaux établissements.

Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, nous sommes réunis aujourd'hui pour débattre d'une proposition de loi importante. Certes, les individus placés en détention détention ont commis des actes répréhensibles. Ces personnes doivent subir une véritable sanction, mais attenter à leur dignité nous semble inadmissible. Fermer les yeux sur des conditions de détention dégradantes n'honore ni notre pays ni notre justice. De nombreux rapports dénoncent à juste titre la surpopulation carcérale, l'impossibilité d'utiliser des sanitaires de manière privée ou la prolifération d'espèces nuisibles dans certains établissements. Si les conditions d'un enfermement digne ne sont pas réunies, l'incarcération risque de perdre tout son sens. Le but de la prison est, bien entendu, de punir, mais elle doit aussi réhabiliter des individus qui, lorsqu'ils auront payé leur dette à la société, devront y être réintégrés. Je tiens à préciser que je ne jette pas la pierre aux personnels de l'administration pénitentiaire, qui essaient de faire au mieux, alors que les conditions ne le permettent pas toujours. Les raisons sont bien connues : personnel en nombre insuffisant, infrastructures vieillissantes et manque de places complexifient inexorablement leur travail. Leurs conditions d'exercice difficiles avaient d'ailleurs été abordées par la commission des lois lors de nos travaux sur l'état des forces de sécurité intérieure.

pour vous faire part de problèmes dont j'ai été témoin lorsque j'ai eu l'occasion de visiter des prisons pour femmes. On parle moins souvent de leurs conditions de détention, mais cela ne signifie pas que leur incarcération se passe sans accroc. accroc. Elles ne représentent que 3,6 % de la population carcérale en France et sont mieux loties que les hommes, certes, en ce qui concerne la surpopulation. Au 1 janvier 2021, on estimait que 2 500 femmes étaient incarcérées pour 2 000 places opérationnelles, mais cette statistique globale cache d'importantes disparités. En effet, certains quartiers pour femmes, comme ceux de Toulouse, Perpignan, Nîmes ou Limoges, sont occupés à plus de 140 %. Ce chiffre peut grimper jusqu'à 170 % à Bordeaux.

Elles sont aussi plus exposées, lors de leur incarcération, aux ruptures de liens familiaux ou conjugaux. Les visites sont plus compliquées pour leurs proches dans la mesure où seuls treize établissements en France accueillent des femmes condamnées à plus de deux ans de prison. Un tel état de fait rend plus difficiles leurs chances de réhabilitation.

dans les premiers mois de leur vie. Environ 60 accouchements auraient lieu chaque année en prison et 95 enfants seraient accueillis chaque année en cellule « mère-enfant Si 29 établissements pénitentiaires sur 191 disposent d'une nurserie, 76 places seulement y sont réservées à des mères avec des enfants. Comme vous le savez peut-être, mes chers collègues, les mères d'enfants de moins de 18 mois peuvent demander à être incarcérées avec leur bébé. la prison de Sequedin, près de Lille, dont je suis ressortie très touchée. Si les mères ont parfois commis des crimes et méritent amplement leur incarcération, leurs enfants, eux, ne sont pas responsables et ils doivent, comme tout être humain, voir leur dignité respectée.

vous rejoignant ainsi, sur ces situations si particulières, et je suis tout à fait ouvert à ce que vous me fassiez part de ce qui vous paraît utile pour améliorer la condition de ces femmes détenues. Monsieur le sénateur Bonhomme, ma réponse à votre intervention sera très rapide, parce que je me félicite de voir que ce texte fait l'objet d'un très large consensus. D'ailleurs, je n'en doutais pas une seconde : comment pourrait-on ne pas être sensible à la surpopulation carcérale et aux conditions indignes

sûr l'honneur de vous en parler, car je sais que la représentation nationale est particulièrement attentive à ces questions. Dans mon esprit, d'ailleurs, il ne s'agit pas d'incarcérer plus, mais d'incarcérer mieux.

discuter ensemble de ces questions plus précisément au travers du projet de loi qui est en cours de finalisation. Enfin, je veux répondre rapidement à M. le sénateur Sueur, qui est particulièrement impliqué sur ces questions. Premièrement, Mme Simonnot,

En réalité, ce sont 6 000 personnes libérées et 6 000 personnes qui ne sont pas entrées en prison. Cette première précision chiffrée est importante. Aujourd'hui, il y a 8 000 détenus de moins qu'en janvier de l'année dernière.

Il serait donc souhaitable que la demande puisse résulter d'une simple audition ou d'un débat. Ce formalisme ne nous apparaît pas nécessaire et peut même constituer un frein important dans certaines situations.

est suffisamment crédible, précise et actuelle, de sorte qu'elle constitue un commencement de preuve de leur caractère indigne, il appartient à la chambre de l'instruction,

l'arrêt qui, en présence d'une description circonstanciée s'arrête au fait qu'elle ne renverrait qu'aux conditions générales de détention dans l'établissement pénitentiaire en cause

Saisie d'une description du demandeur, qui évoquait une cellule infestée de punaises et de cafards, l'absence de chaise, la saleté la saleté repoussante des douches et le sous-dimensionnement de la cour de promenade, la chambre de l'instruction devait en apprécier le caractère précis, crédible et actuel, sans s'arrêter au fait que cette description ne renverrait qu'aux conditions générales de détention à la maison d'arrêt de Fresnes, ni exiger du demandeur qu'il démontre le caractère indigne de ses conditions personnelles de détention. » J'en conclus que les amendements

que la requête soit recevable dès lors qu'il y a de simples indices, en vous fondant sur l'arrêt du 25 novembre 2020 de la Cour de cassation. Permettez-moi de vous dire, puisque vous l'invoquez régulièrement et que vous allez le faire encore,

pourrait présenter de simples indices de conditions de détention indignes. Pour ma part, je suis attaché à l'équilibre de la proposition de

selon des critères assez simples et ne reposant que sur des indices, à faire libérer leurs clients. Il me paraît donc important que les demandes soient un minimum étayées.

il y a aussi une réalité : les juges de l'application des peines et les juges des libertés et de la détention ont beaucoup de travail.

À cet égard, je dois quand même revenir sur les propos de M. le rapporteur. Je vois bien ce qu'il dit : « Ce texte nous fait peur,

or il ne me paraît pas déraisonnable de laisser au moins trois jours à l'administration pénitentiaire pour rassembler des éléments et préparer sa réponse. Si l'on adoptait cet amendement,

S'il est écrit dans la loi que l'administration pénitentiaire a dix jours pour statuer, le juge ne va pas en conclure, comme le fait M. Frassa en vertu d'une logique qui lui est propre,

vise à préciser- on m'a affirmé que c'était implicite, mais écrivons-le explicitement -que le détenu peut agir seul, sur sa propre initiative, et être auditionné seul sans que la présence d'un avocat soit nécessaire. Chacun comprendra ce que cela veut dire, c'est d'une clarté limpide, et je ne vois pas pourquoi il y aurait des oppositions à cet amendement. Quel est l'avis de la commission ? Là, monsieur Sueur, j'avoue que c'est un amendement pour faire un amendement

je vous ai répondu que le texte ne demandait pas la lune, si vous me permettez cette familiarité ; or voilà que maintenant il faudrait préciser que le détenu peut agir seul, alors que l'avocat n'a pas été prévu ! Je suis

Nous y demandons que tous les documents, pièces et informations obtenus à l'occasion de ce contrôle soient versés au dossier, adressés aux parties et débattus contradictoirement.

Cet amendement vise donc à renforcer l'information des parties et leur présence dans la procédure afin d'assurer un strict respect des droits de la défense. Toutes les vérifications et observations recueillies par le juge auprès de l'administration pénitentiaire

: il y est proposé que tous les documents et informations obtenus par le juge soient transmis aux parties et débattus contradictoirement. Nous ne sommes pas ici dans le cadre d'une information judiciaire. Les exigences procédurales doivent être compatibles avec le prononcé d'une décision que l'on veut rapide. C'est bien l'esprit même de cette proposition de loi, qui prévoit déjà que toutes les parties pourront faire connaître leurs observations et que le détenu lui-même pourra demander à être entendu par le juge avant qu'il ne rende sa décision, ce qui garantit à mon sens le respect du principe du contradictoire. Il ne me paraît cependant pas raisonnable d'aller au-delà ; l'avis de

garde des sceaux. Je suis très flatté, monsieur le sénateur Sueur : si je vous comprends bien, votre amendement est devenu totalement inutile après mon intervention.

Néanmoins, c'est une réalité humaine insoutenable et, lorsque se produisent des faits de cet ordre, il n'est pas exorbitant de demander que les délais soient raccourcis. raccourcis. L'objet de cet amendement est justement de réduire le délai laissé par le juge à l'administration pénitentiaire pour mettre fin, par tout moyen, à ces conditions de détention. Dans la proposition de loi, le délai entre le moment où le juge reçoit

Il faut s'assurer que toute action de l'administration n'ait pas d'impact sur la requête. Nous proposons donc de réduire ce délai à moins de dix jours.

le juge ne peut pas enjoindre à l'administration pénitentiaire de prendre des mesures déterminées pour mettre fin aux conditions indignes de détention.

En effet, la réserve formulée dans la proposition de loi est problématique, puisqu'elle prive le magistrat de pouvoir intervenir réellement sur les conditions de détention et laisse l'administration- pour laquelle j'ai le plus grand respect -seul maître,

pour l'effectivité de ce nouveau recours. L'amendement vise un objectif d'intérêt général- la sauvegarde de la dignité humaine -, qui

que l'alinéa 3 de l'article 803-8 de la proposition de loi comprend déjà une injonction à l'administration de faire connaître, dans un délai déterminé, les mesures

de la seule compétence de la juridiction administrative. Il est certes loisible au législateur, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de constituer des blocs de compétences pour éviter que la dualité de juridiction soit source de désordres procéduraux dans un domaine déterminé.

amendement. Avec le dispositif actuel, c'est en premier lieu à l'administration pénitentiaire d'agir. Il lui suffit donc de proposer un transfert pour neutraliser la perspective d'une libération, choix qui reste possible possible dès lors que le juge en décide, en vertu même de la présente proposition de loi. Or cette solution n'est pas satisfaisante et risque de dissuader la personne détenue d'effectuer un recours. Les personnes

prisons. Une fois le requérant transféré, il est probable qu'un autre prendra sa place- sauf à faire tous les travaux de construction, de reconstruction, de canalisation, chers à M. le garde des sceaux

présente un taux d'occupation plus satisfaisant, il est parfaitement légitime que l'administration pénitentiaire procède à un transfèrement afin d'améliorer les conditions de détention.

Madame Benbassa, le maintien des liens familiaux est une préoccupation constante de l'administration pénitentiaire. La proposition de loi y apporte une garantie importante, puisqu'elle précise qu'un condamné peut légitimement refuser un transfèrement au motif qu'il aurait porté atteinte excessive à sa vie familiale. La situation des personnes placées en détention provisoire est, quant à elle, différente, car il faut, dans ce cas, tenir compte des nécessités de l'enquête

le réexpliquer. Nous sommes contre la décision de transfèrement par l'administration pénitentiaire avant la décision du juge. Est-ce clair ? est-ce que cela signifie que nous sommes contre le transfèrement ? Nous ne sommes pas du tout contre le transfèrement : nous sommes pour que le transfèrement ait lieu, le cas échéant, après saisine et décision du juge.

et où les transferts s'avèrent illusoires, font obstacle à ce que l'utilisation du référé-liberté offre aux personnes détenues la possibilité en pratique de faire cesser pleinement et immédiatement

Le texte élaboré par la commission prend déjà en compte la dimension des liens familiaux, et la procédure proposée est respectueuse des droits de la défense. Concernant les aspects sanitaires et sociaux, il serait surprenant que le détenu qui souffre de conditions de détention indignes

proposer une notion d'« examen approfondi de la situation familiale et sociale » du détenu, qui est très vague. Quels seraient alors les critères appliqués par le juge ? Un détenu dont la situation sociale est très difficile ne pourrait-il bénéficier d'un transfèrement, ou serait-il au contraire prioritaire ?

l'avis de la commission ?

nous proposons de restreindre la visioconférence aux cas de force majeure.

le détenu ne bénéficiera pas de la mesure de libération décidée par le juge en attendant que l'appel soit jugé. Il est donc dans l'intérêt du détenu que le jugement intervienne rapidement. C'est pourquoi il serait malvenu de supprimer le délai de quinze jours : avis défavorable. Quel est l'avis Vous avez raison, monsieur Sueur, il faut être patient. Pour ne rien vous cacher, j'ai le sentiment ce soir de l'être particulièrement. Je

Je ne vous étonnerai donc pas en vous disant que je suis totalement défavorable à votre amendement.

aux différentes condamnations de la Cour européenne des droits de l'homme. Dans son arrêt du 30 janvier 2020, que j'ai la Cour européenne des droits de l'homme pointait un problème structurel en matière de surpopulation carcérale en France et exigeait l'adoption de mesures générales visant à supprimer le surpeuplement et à améliorer les conditions matérielles de détention.

L'inflation carcérale que connaît la France depuis plusieurs décennies est avant tout le fruit des politiques pénales antérieures. Je connais la diversité des gouvernements qui se sont succédé, et je ne ferai aucun simplisme à cet égard.

Je finirai en mentionnant le rapport parlementaire d'information sur les moyens de lutte contre la surpopulation carcérale, présenté par Dominique Raimbourg et Sébastien Huyghe, en 2013. Ce serait une bonne lecture, car ses auteurs ont pris le risque de formuler des propositions qui n'allaient pas de soi, mais qu'il serait peut-être bon de prendre en compte.

Gouvernement pourrait nous donner des indications sur la manière dont il envisage l'évolution du taux d'occupation carcérale dans les prochains mois et dans les prochaines années. L'ouverture de nouvelles places de prison devrait contribuer à le faire baisser, de même que la mise en oeuvre de la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice,

Le Gouvernement, par votre voix, pourrait donc utilement nous éclairer sur la stratégie qu'il compte suivre en matière de gestion de la population carcérale.

Certains ont pensé qu'il s'agissait d'avancer vers les aménagements de peine et d'autres d'être plus restrictif. Il est évident qu'être plus restrictif ne permettra pas de lutter contre la surpopulation

La juridiction de l'application des peines peut aménager les peines d'emprisonnement ferme en prononçant l'une des mesures suivantes : libération conditionnelle, suspension de peine pour raisons médicales, semi-liberté, placement à l'extérieur ou placement sous surveillance électronique. Des permissions de sortie peuvent également être accordées sous certaines conditions. Le tribunal correctionnel peut aussi décider, dès la condamnation, que la peine d'emprisonnement fera l'objet d'un aménagement. Ce rapport, qui n'existera pas lequel nous appelons l'attention du Gouvernement, permettrait d'y voir clair et d'évaluer l'effet de ces aménagements de peine sur la nécessaire lutte contre la surpopulation pénitentiaire.

pourrait faire évoluer les dispositions relatives à la libération sous contrainte déjà modifiées par la loi de programmation du 23 mars 2019. À cette occasion, nous aurons sans doute le plaisir d'entendre le garde des

d'autant que, je le répète, tous les chiffres sont publiés régulièrement, vous en prenez connaissance et, comme vous connaissez bien la matière, vous savez parfaitement quelle est l'action du Gouvernement.

Ainsi, nous aurions pu dire que la proposition de loi tend « à assurer l'effectivité du droit au respect de la dignité en détention ». Comme il n'en est rien, hélas, nous retirons cet amendement.

Nous avons cité nos sources : Mme la Contrôleure générale des lieux de privation de liberté, l'Observatoire international des prisons, l'interprétation qui nous paraît claire de l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme,

de l'ensemble de ces auditions et de ces contacts, il est apparu que ce texte devait être précisé et amélioré afin que le droit à saisir le juge judiciaire pour les détenus en situation d'indignité soit effectif. Nous avons même déposé une proposition de loi qui rassemblait ces différentes modifications. Je dois dire, pour être tout à fait juste, l'une de nos propositions a été retenue en commission. Alors que le texte prévoyait initialement que le juge pouvait auditionner la personne,

pas. Nous nous abstiendrons au motif que nos différentes propositions- elles ne sont pas seulement les nôtres -n'ont malheureusement pas pu être prises en compte. Toutefois, nous gardons l'espérance- il faut toujours avoir une lueur d'espoir -qu'elles pourraient l'être par l'Assemblée nationale. Personne ne